La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 21 mars 2019 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Marcel-Pierre Cléach, qui fut sénateur de la Sarthe de 1995 à 2014.

Cette aide ne saurait ainsi être attribuée qu'en l'absence d'alternative par les transports en commun. Il s'agit donc d'encourager prioritairement les transports collectifs, et non individuels.

congestion ou la pollution de l'air- nous avons eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Toutefois, le développement du covoiturage de courte distance se heurte à certains obstacles, en particulier le faible intérêt économique qu'y trouvent les covoitureurs,

Sur le territoire francilien, par exemple, où l'offre de transports publics est dense, on voit bien à quel point le développement du covoiturage permettrait de réduire les embouteillages et la pollution de l'air. L'expérimentation « Tous ensemble pour le covoiturage », menée

de ceux-ci. Dans beaucoup de territoires, il n'existe pas d'alternative à la voiture individuelle ; dans ces territoires, il est évidemment très important de permettre aux autorités organisatrices d'encourager le développement du covoiturage,

est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote. Je trouve ces deux amendements très intéressants. Madame la ministre, vous venez de préciser que le covoiturage est une solution pertinente là où il n'y a que très peu de transports en commun disponibles. Il n'empêche

Par cet amendement de bon sens, nous demandons simplement, au regard des nouvelles compétences des autorités organisatrices en matière de covoiturage, que la

? En matière de développement des mobilités partagées, comme dans d'autres domaines, d'ailleurs, l'intervention publique est utile lorsqu'elle vient pallier les carences du secteur privé et répondre à un besoin qui n'est pas satisfait. Si les besoins sont déjà satisfaits, je ne vois pas en quoi un acteur public serait fondé à venir

il paraît effectivement pertinent que les autorités organisatrices interviennent dès lors qu'il existe une carence de l'offre privée. Il n'y a aucun intérêt à mobiliser des financements publics si des acteurs privés répondent déjà aux besoins de ceux qui veulent pouvoir recourir au covoiturage.

d'une part, de permettre aux communes d'Île-de-France de créer des plateformes de covoiturage, dans une logique de subsidiarité avec Île-de-France Mobilités, dans le cas où l'établissement

d'autre part, d'encadrer les conditions de délivrance du signe distinctif de covoiturage. L'article 15 prévoit la possibilité de créer des emplacements de stationnement réservés aux véhicules porteurs d'un signe distinctif de covoiturage, mais les conditions de délivrance de ce signe ne sont pas précisées. Il s'agirait donc de préciser que ces conditions de délivrance sont les mêmes que celles des signes distinctifs relatifs au label « autopartage

? Je pourrais faire une réponse courte en disant que « mobilité » rime avec « lisibilité » et avec « visibilité ». Mais je vais détailler quelque peu mon avis. En matière de mobilités, la situation de la région francilienne est en effet atypique, compte tenu de la présence d'une autorité organisatrice unique, Île-de-France Mobilités. La densité de la démographie et des flux de personnes sur ce territoire justifie que la question de la mobilité soit appréciée à une échelle large. Permettre à chaque commune du territoire francilien de créer sa propre plateforme de covoiturage ou son propre signe distinctif de covoiturage- je réitère d'ailleurs mon propos précédent sur l'utilisation de l'argent public -, alors même que l'enjeu de la mobilité dépasse de loin le cadre communal, paraît hasardeux et source potentielle de complexité pour les automobilistes, en cas de multiplication des labellisations « covoiturage ». Avis défavorable,

Donner cette possibilité à chaque commune pourrait, comme vient de le dire M. le rapporteur, être source de complexité et faire perdre en lisibilité. Au demeurant, cela créerait une différence avec la situation des autres régions,

mobilités. Il s'agit d'offrir la possibilité aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale de créer des zones à trafic limité sur tout ou partie de leur territoire lorsqu'un plan de mobilité a été adopté ou est en cours d'élaboration ou de révision. De telles zones permettent d'assurer la tranquillité, la sécurité et la sûreté des voies publiques ; elles ont aussi pour vocation de favoriser la lutte contre la pollution atmosphérique. Ces zones sont dites à trafic limité en ce que certains véhicules sont autorisés à y circuler après avoir obtenu une autorisation de circulation. Le principe est bien de pacifier certains quartiers en éliminant la circulation de transit au sein d'un périmètre donné, sans toutefois empêcher les riverains et un certain nombre d'ayants droit de circuler ou de stationner, et sans modifier les règles de priorité et d'usage de la chaussée. L'existence de ces zones peut ne valoir que durant certaines périodes. Il est nécessaire de souligner que de telles zones de circulation restreinte existent déjà dans d'autres pays européens tels que l'Allemagne et l'Italie ; il serait intéressant que la France leur emboîte le pas. Quel est l'avis de la commission

: mettre en place des zones à trafic limité, c'est-à-dire des zones qui seraient uniquement accessibles à certaines catégories de véhicules, voire à des véhicules précis, autorisés. À cet effet, vous reprenez la procédure prévue pour les zones à faible émission, dispositif très contraignant assorti d'un processus d'études et de consultation lui-même contraignant. Comme l'a évoqué M. le rapporteur, les dispositions des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et la partie réglementaire du code de la route permettent déjà la création, dans un cadre juridique souple, d'aires piétonnes et de zones à trafic limité. C'est d'ailleurs ce qui a été fait par la ville de Nantes. Cependant, je suis sensible à ce que notre droit soit lisible. J'ai donc demandé à mes services d'identifier par quelles voies les possibilités du droit existant en la matière pourraient être rendues plus explicites

En commission, nous avons en effet souhaité permettre aux maires de créer des voies de circulation ou des emplacements de stationnement réservés, non pas seulement pour les véhicules à très faibles émissions, qui ne concernent qu'une très faible part des véhicules en circulation, mais, plus généralement, pour certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques. Il s'agit donc de donner de la souplesse aux maires

amendement vise par ailleurs à introduire la possibilité pour le maire de ne pas autoriser, sur ces voies réservées, les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes, pour des raisons de sécurité routière. J'ajoute que le maire sera libre de choisir quel véhicule il autorise parmi les catégories autorisées et en leur sein.

de permettre au transport public de bénéficier d'un avantage par rapport à l'autosolisme- je parle en termes de vitesse commerciale. Afin que l'impact sur le transport public et sur la congestion reste limité de la répartition des compétences, la charge revenant soit à l'autorité organisatrice de la mobilité, soit au maire, il paraît nécessaire de s'assurer de l'avis conforme de l'autorité organisatrice de la mobilité pour ne pas se retrouver avec des sites propres saturés, comme j'ai pu le constater à Milan il y a quelques années.

Comme Didier Mandelli a davantage évoqué les véhicules de fort tonnage, je veux m'assurer qu'il n'y a pas méprise, et que l'ensemble des véhicules

pour certaines catégories de véhicules sur les voies dont ils ont la gestion. C'est le principe qui nous guide depuis le début de l'examen de ce texte : laissons les maires décider. Prévoir que les maires sont obligés d'avoir l'accord des autorités organisatrices de la mobilité avant de pouvoir créer de telles voies réservées constituerait une restriction importante à leur pouvoir de police de la circulation,

Mais je pense qu'il serait gênant d'introduire un avis conforme de l'autorité organisatrice sur une prérogative qui dépend du pouvoir de police, ce qui pourrait freiner le développement de ces voies réservées.

les motorisations prévues sont les véhicules électriques, à hydrogène, les hybrides rechargeables, les hybrides non rechargeables et les véhicules à air comprimé. Les carburants alternatifs, comme le gaz de méthanisation, ne figurent pas sur la liste.

l'amendement n° 879. Cet amendement a pour objet de permettre aux communes de créer des espaces de logistiques urbains pour fluidifier les livraisons sur leur territoire. Le développement du commerce électronique et des livraisons individuelles a entraîné la multiplication de la circulation des poids lourds en ville. Cette circulation est source de nombreuses nuisances : congestion, pollution de l'air, bruit, dégradation des chaussées ... Il est indispensable de développer de nouvelles solutions pour permettre d'assurer le dernier kilomètre de livraison avec des véhicules propres et adaptés aux centres urbains. C'est tout l'objet de ces espaces logistiques, pouvant accueillir des conteneurs ou autres moyens de stockage à même de servir d'interface en accueillant la cargaison d'un poids lourd avant sa ventilation progressive pour être livrée en plusieurs endroits par des véhicules légers. Ces espaces peuvent être créés hors voirie, mais leur réalisation bute sur des coûts importants et une disponibilité foncière rare. Pour pallier cette difficulté, il est donc souhaitable d'utiliser l'espace public pour y créer des espaces logistiques. Pour en permettre le respect par les autres usagers, ils doivent pouvoir faire l'objet d'une réservation au titre des pouvoirs de police du maire, sous réserve d'une mise en concurrence préalable en vue d'obtention d'une convention d'occupation du domaine public. Cette réservation peut être temporaire et utilisée à certains horaires à des fins de stationnement. Il serait également pertinent, à l'occasion de la modification de l'article, de donner un fondement législatif à la création de voies cyclables, et d'emplacements de stationnement réservés pour les cycles, engins de déplacement personnel, cyclomoteurs ou motocyclettes. La

Ces amendements visent à aller beaucoup plus loin, en leur permettant de créer des espaces logistiques sur la voie publique pour faciliter les livraisons par des véhicules peu polluants. Mais créer de tels espaces, dont les dimensions seraient potentiellement importantes, sur la voie publique conduirait à encombrer les voies de circulation.

fois de créer des espaces de logistique urbaine et de réserver des espaces pour le déplacement des deux-roues et engins de déplacement personnel.

Sur les deux-roues, les textes en vigueur permettent déjà de réserver des voies de circulation aux cycles et des emplacements de stationnement ciblés à cet effet. La question des règles applicables aux engins de déplacement personnel- c'est un véritable sujet pour les piétons qui veulent se déplacer sereinement sur les trottoirs

La problématique existe déjà sur Paris, mais aussi dans d'autres villes, avec la dépose de conteneurs, qui permettent ensuite de faire le lien avec des véhicules plus légers. C'est cette dépose qui pose problème. Comme cela

la congestion des centres-villes est un fléau moderne. Elle détériore le cadre de vie par ses nuisances sonores et son invasion-colonisation de l'espace. Plus grave, elle nuit à la santé des habitants en dégradant la qualité de l'air. De plus en plus d'élus locaux cherchent à se réapproprier leur centre-ville en limitant la place de la voiture, qui, rappelons-le, occupe jusqu'à la moitié de l'espace public disponible en ville. Il nous paraît donc nécessaire d'augmenter l'arsenal juridique de solutions à leur disposition.

permettrait de pacifier certains quartiers en éliminant la circulation de transit au sein d'un périmètre donné, sans toutefois empêcher les riverains et un certain nombre d'ayants droit de circuler à une vitesse réduite à 20 kilomètres par heure ou de stationner, sans modifier les règles de priorité et d'usage de la chaussée.

est satisfait par le droit existant, qui permet déjà aux maires de créer des aires piétonnes et des zones à trafic limité. L'article R. 110-2 du code de la route mentionne expressément les aires piétonnes. Les zones à trafic limité, au sein desquelles la circulation est interdite sauf pour certaines catégories de véhicules, peuvent également être mises en place par les maires, dans le cadre de leur pouvoir de police de la circulation. Une telle zone a d'ailleurs été mise en place par la ville de Nantes. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas besoin de dispositions législatives supplémentaires.

d'éviter les contentieux, tout en facilitant les déplacements et la circulation, donc la mobilité, sur ces espaces, avec les techniques les

d'ores et déjà d'un pouvoir de police générale sur les routes nationales et les autoroutes. À ce titre, ils peuvent réserver la circulation à certains usagers sur les autoroutes et les routes express. Au demeurant, c'est déjà le cas. Des voies réservées ont été créées sur certaines autoroutes.

en service sur l'A 12, l'A 10, l'A 6a, l'A 1 en Île-de-France. Il y a des projets sur la RN 118 et sur l'autoroute A 3. S'agissant des bandes d'arrêt d'urgence, il y a déjà des projets en service sur l'A 48 à Grenoble,

Quel est l'avis du Gouvernement ? L'avis du Gouvernement reste défavorable. On est en train d'empiler des règles de droit, en renvoyant à des décrets,

à permettre sous condition aux maires, au titre de leur pouvoir de police en matière de circulation, de demander au préfet une application différenciée des limitations de vitesse, selon leur dangerosité, de routes ou de portions de routes relevant de leur propre domaine.

Nous nous situons en dehors des débats que nous avons déjà pu avoir sur la règle du 80 kilomètres par heure. Cet amendement vise à offrir une marge de manoeuvre supplémentaire aux maires dans la régulation de la vitesse sur le territoire de la commune, où la vitesse maximale autorisée est, comme vous le savez, fixée à 50 kilomètres Or, dans un nombre significatif de communes, il est courant d'observer des portions de voies situées en dehors des zones résidentielles, où il pourrait être techniquement possible de rouler à des vitesses supérieures sans dégrader la sécurité routière. C'est notamment le cas de certaines voies assurant la transition avec les routes nationales et départementales, où il est courant de voir des automobilistes verbalisés alors qu'ils pensaient de bonne foi se situer en dehors de la zone réglementée par la commune. Cette situation est souvent rendue encore plus complexe par le caractère peu clair de la signalisation sur certaines voies. Pour cette raison, il pourrait être pertinent d'autoriser le maire à édicter des vitesses maximales supérieures sur ce genre de portions. Afin de prévenir les éventuels abus, une telle mesure serait soumise avant son application à l'avis conforme du représentant de l'État, qui pourra au besoin consulter la commission départementale de la sécurité routière sur l'opportunité de relever les vitesses maximales. Quel

des vitesses maximales autorisées par le code de la route pour les adapter en fonction de la dangerosité des routes. Si le maire ou le président de département identifient un tronçon dangereux sur le réseau routier national pour lequel la vitesse nécessite selon eux d'être abaissée, ils peuvent saisir le préfet de demandes en ce sens sans qu'il soit besoin d'une disposition législative. Avec une telle rédaction, ces amendements ne changent rien à la législation actuelle. En revanche,

eu égard aux nécessités en matière de protection de l'environnement, de réserver des emplacements de stationnement pour les véhicules propres ou à faibles émissions dans l'atmosphère de CO2 ou de polluants.

autant quand on met en place des zones à faibles émissions, il faut évidemment prendre en compte la nécessité de laisser ces zones accessibles à tout un chacun, autant quand on est en train de donner des avantages à l'usage, ces avantages à l'usage, pour être efficaces, doivent être réservés aux véhicules

est à M. Alain Duran. Cet amendement vise à permettre sous condition aux conseils départementaux de procéder à une application différenciée des limitations de vitesse selon la dangerosité des routes du domaine départemental, en modifiant

son rôle n'est pas de faire obstruction au travail du Gouvernement ou du Président de la République

sur la question de l'application du 80 kilomètres par heure, cet amendement vise à rendre l'abaissement de la limitation moins rigide en offrant des marges de manoeuvre au préfet et au président du conseil départemental. Alors que la gestion des vitesses maximales autorisées est au coeur de la problématique de nombreux territoires enclavés ou périphériques, selon l'expression consacrée, il est critiquable d'avoir fait le choix d'une application uniforme de la règle du 80 kilomètres par heure sur l'ensemble du territoire national. Ce choix est d'autant plus problématique que son efficience réelle en matière de sécurité routière est discutable. Nos voisins allemands appliquent, par exemple, des vitesses maximales supérieures à celles de la France, tout en comptant moins de morts chaque année sur les routes. La sécurité routière est bien sûr un élément fondamental, mais elle ne peut pas être le critère unique en matière de délimitation de vitesse. L'enclavement des territoires en est, par exemple, un autre tout aussi fondamental. En conséquence, cet amendement vise à permettre au président du conseil départemental et au préfet de rehausser les vitesses maximales sur les routes départementales et nationales, après

Duran. Cet amendement vise à permettre sous condition aux conseils départementaux de demander au préfet une application différenciée des limitations de vitesse, selon leur dangerosité, de routes ou de portions de routes relevant du domaine routier national.

notamment au regard de l'objectif du Gouvernement de sauver quatre cents vies supplémentaires par an. Même si nous avons conscience qu'il est toujours complexe d'effectuer un premier bilan après un an, nous pensons que les éléments qui ont pu remonter jusqu'ici sont suffisants pour envisager une première approche globale. De plus, nous gardons également en tête les déclarations du Président de la République sur ce sujet, lequel s'est engagé à moduler la mesure selon les besoins, voire à l'abandonner dans le cas où les résultats ne seraient pas suffisants.

Le Gouvernement s'est engagé, lors de la mise en place de cette mesure, à ce qu'elle fasse l'objet d'une évaluation deux ans après son entrée en vigueur, c'est-à-dire au 1 juillet 2020, afin d'étudier ses effets sur l'accidentalité. Cet amendement va dans ce sens, mais vise à avancer la date du rapport, qui serait remis six mois après la promulgation de la loi, c'est-à-dire vraisemblablement vers le mois de janvier 2020. Mesurer l'effet sur l'accidentalité des 80 kilomètres par heure nécessite un temps statistique suffisamment long ; je ne suis pas sûr qu'il soit opportun d'avancer la remise du rapport de quelques mois.

présenter un bilan du décret du 15 juin 2018 et de l'adresser à l'ensemble des gestionnaires de voirie pour bien mesurer les résultats de l'accidentalité et de la mortalité routière à la suite de l'abaissement des vitesses maximales.

libellé : La parole est à Mme Michèle Vullien. L'article 15, inséré en commission, vise à prévoir la possibilité pour les collectivités de moduler le tarif des redevances de stationnement pour les personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale, et pour celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite. du code de l'action sociale et des familles prévoit déjà la gratuité du stationnement pour les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». La mention d'une tarification spécifique en faveur des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite viendrait donc complexifier, voire insécuriser, le système actuel dans lequel des personnes en situation de handicap bénéficient déjà de l'accès gratuit au stationnement. L'amendement vise à recentrer la tarification solidaire au profit des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, en tenant compte de leur revenu ou de leur statut, dans un motif d'égalité d'accès à la mobilité. Quel

peuvent l'être selon deux modalités. Soit l'avis de paiement du FPS est déposé sur le pare-brise du véhicule concerné au moment du contrôle, soit il est envoyé par voie postale au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation. Dans ce deuxième cas, les collectivités ont obligatoirement recours aux services de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, l'ANTAI, seule habilitée à accéder aux fichiers où sont consignées les informations personnelles- nom, adresse -des propriétaires des véhicules. ayant recours aux services de l'ANTAI ont toutes signé avec cette dernière une convention d'une durée de trois ans, qui arrive à échéance au 31 décembre 2020. Afin de renforcer la décentralisation de la gestion du stationnement par les collectivités et de leur donner davantage de latitude dans la mise en oeuvre de leur politique, le présent amendement vise à ouvrir l'accès au système d'immatriculation des véhicules à toutes les collectivités chargées de collecter la redevance de stationnement sur voirie. Quel

traitement automatisé des infractions, ce qui simplifierait les démarches. Toutefois, permettre à tous les agents de surveillance de la voie publique d'accéder au système d'immatriculation des véhicules pourrait alourdir la gestion de ce fichier et nécessiterait un encadrement pour assurer la protection des données

chargées de collecter les redevances de stationnement sur voirie. Il vise donc à supprimer le rôle de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions dans l'envoi de l'avis de forfait post-stationnement.

taille très inégale, et en sécurisant le traitement des données personnelles. En 2018, plus de 8 millions de forfaits post-stationnement ont été traités pour le compte de plus de 500 collectivités ayant signé une convention avec l'ANTAI. L'ouverture du système d'immatriculation des véhicules aux collectivités mettant en oeuvre la décentralisation du stationnement payant aurait pour effet d'augmenter significativement le nombre d'acteurs habilités à consulter ce fichier, ce qui pose

Elles peuvent également choisir de transmettre cette mission à leur autorité organisatrice de la mobilité, c'est-à-dire, le plus souvent, à leur établissement public de coopération intercommunale, ou EPCI, à fiscalité propre. En Île-de-France, du fait de la spécificité de l'organisation institutionnelle de cette région, c'est Île-de-France Mobilités qui est ciblé comme potentiel destinataire de cette mission. Le présent amendement vise à modifier ces dispositions, en ajoutant les EPCI à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux dans la liste des collectivités que les communes franciliennes peuvent identifier comme destinataires de la capacité d'instaurer la redevance de stationnement. Les conditions requises pour que ce transfert soit effectif sont les mêmes que celles qui sont retenues dans le cadre du transfert communes-EPCI hors Île-de-France. Quel La mise en place d'une redevance de stationnement peut être décidée par les communes ou par les EPCI, qui sont compétents en matière d'organisation des mobilités, après accord des communes. Dans la région francilienne, c'est l'autorité organisatrice Île-de-France Mobilités qui est susceptible de bénéficier de ce transfert de compétence pour mettre en place des redevances de stationnement. Cet amendement vise à permettre aux EPCI franciliens et aux établissements publics territoriaux, qui ne sont pas compétents en matière de mobilité, de pouvoir bénéficier d'un tel transfert de compétence. Cet amendement tend à offrir de la souplesse, et c'est ce que nous recherchons. Voilà pourquoi la commission est favorable à son adoption. à son adoption. Quel est l'avis du Gouvernement ? Effectivement, en dehors de l'Île-de-France, les communes peuvent décider de permettre à leur autorité organisatrice de mobilité, c'est-à-dire le plus souvent à leur établissement public de coopération intercommunale, d'instaurer une redevance de stationnement payant. En Île-de-France, c'est Île-de-France Mobilités qui est identifié comme collectivité susceptible de bénéficier de ce transfert de mission. L'amendement vise à permettre, dans cette région, aux EPCI à fiscalité propre et aux établissements publics territoriaux d'instaurer cette redevance de stationnement, après accord d'Île-de-France Mobilités. Il est en effet souhaitable de permettre une plus grande proximité,

Aujourd'hui, les professionnels de la location de véhicules rencontrent des difficultés pour percevoir le remboursement par le locataire du forfait post-stationnement, c'est-à-dire l'amende. Ainsi, le système actuel a des conséquences considérables sur la pérennité économique du secteur, car le montant de ces droits est parfois bien supérieur au bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Dans votre réponse à ma question écrite, vous m'aviez précisé, madame la ministre, qu'il s'agissait désormais d'un sujet de droit civil contractuel entre le propriétaire du véhicule, seul redevable envers l'administration, et la personne à laquelle il confie son véhicule et qui est contractuellement responsable de son bon usage. Vous renvoyiez à l'adaptation des conditions générales de vente, avec de nouvelles clauses ne pouvant être considérées comme des clauses abusives. Afin de simplifier le système sans pour autant remettre en cause la construction juridique de la réforme du stationnement payant, je vous propose d'introduire une possibilité de désignation ouverte aux loueurs, sur le modèle des dispositions applicables aux amendes des radars, et ainsi de transmettre automatiquement le paiement de la redevance d'occupation du domaine public, due actuellement par le titulaire du certificat d'immatriculation.

de désigner le locataire responsable, elles doivent désormais s'acquitter d'abord d'un forfait post-stationnement, avant de se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme.

Ces professionnels apportent pourtant une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, en offrant une alternative à la possession d'un véhicule, et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile. Nous ne pouvons donc laisser perdurer une telle injustice, une telle désincitation à leur égard. Aussi, en ciblant les professionnels de l'automobile, cet amendement a pour dessein de leur permettre de désigner leurs clients responsables du non-paiement de stationnement, afin non seulement de rétablir une égalité de traitement vis-à-vis des loueurs de longue durée, mais également de mettre fin au sentiment d'impunité des clients qui ne paient pas, volontairement, leur forfait post-stationnement. La parole

a modifié les conditions d'application du forfait post-stationnement pour les automobilistes qui sont en infraction au regard des règles de stationnement. En l'absence de paiement ou en cas de paiement insuffisant, le titulaire du certificat d'immatriculation

cette préoccupation ne doit pas conduire à revoir les principes mêmes de la réforme du stationnement payant, entrée en vigueur le 1 janvier 2018, et qui prévoit un système de redevance construit autour d'un redevable unique

n'ont pas nécessairement encore trouvé leurs marques. Pour autant, il n'est pas souhaitable de revenir sur la philosophie selon laquelle le forfait post-stationnement est payé par le titulaire du certificat d'immatriculation.

aux agents de surveillance de la Ville de Paris, de manière transitoire, avant la mise en oeuvre effective de la police municipale parisienne. Il est également proposé d'étendre le contrôle aux aires piétonnes et aux voies cyclables afin d'en contrôler mieux l'usage, car nous sommes confrontés à de nombreuses incivilités. Il s'agit de garantir, notamment à Paris, un plus grand respect des voies réservées à un certain nombre de véhicules et de permettre une verbalisation plus efficace et plus étendue.

afin de sanctionner plus facilement les conducteurs qui empruntent des voies réservées. Ce dispositif va mêler images de vidéosurveillance, accès à certains fichiers, et même capteurs capables de détecter le nombre de passagers à bord d'un véhicule. Ainsi, afin d'identifier les contrevenants, les numéros de plaque d'immatriculation des véhicules

des moyens techniques actuels, la mise en place de tels procédés, en particulier pour le contrôle des zones à faibles émissions, les ZFE, pourrait revenir à autoriser une surveillance massive des personnes en circulation, et ce en contradiction avec la liberté d'aller et venir anonymement. Sans doute est-ce pour cela que le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi : « Le recueil systématique des photographies de plaques d'immatriculation des véhicules circulant sur l'ensemble des voies réservées sur le territoire national et, par conséquent, de leurs conducteurs et passagers, susceptibles ainsi d'être identifiés, est de nature à permettre la saisie sur une grande échelle de données personnelles, relatives au déplacement des individus

conducteur doit rester identifiable. L'alinéa 8 de l'article 16 encadre strictement les conditions dans lesquelles les données permettant l'identification du conducteur du véhicule sont communiquées. S'il est préférable de ne pouvoir accéder qu'à l'image du conducteur, les technologies actuelles ne permettent pas encore de manière fiable de procéder à la distinction entre le conducteur et les autres passagers du véhicule.

permettant de protéger au maximum les libertés publiques. C'est pourquoi je propose de modifier la phrase concernant le traitement des images collectées, tout en précisant que les occupants ne doivent pas être identifiables, sauf dans les cas strictement nécessaires aux procédures de traitement des infractions et réclamations.

Les modalités de consultation des fichiers et de traitement des données personnelles prévues à l'article 16 sont limitées et proportionnées à la finalité recherchée. Je rappelle par ailleurs que les actes réglementaires d'application de ces dispositions seront soumis à l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, et que la mise en place des dispositifs de contrôle devra, à chaque fois,

en commission, ainsi qu'avec ma collègue Françoise Gatel, rapporteur pour avis de la commission des lois, prévoir que les données issues des contrôles automatiques des voies réservées fassent l'objet d'un traitement permettant de masquer de manière irréversible l'identité des passagers et des tiers des véhicules. Il s'agit ainsi de renforcer la protection des données personnelles dans le cadre de la mise en place de ces dispositifs de contrôle. D'après les informations qui nous ont été transmises, lesquelles ont

inquiété du « recueil systématique des photographies de plaques d'immatriculation des véhicules ». La CNIL a également recommandé des garanties supplémentaires. l'initiative des rapporteurs, nous l'avons évoqué, un masquage immédiat et irréversible des images permettant l'identification des passagers et des tiers parce que celle du conducteur suffit que cela ne remet pas en cause l'efficacité du dispositif. Dans votre amendement, madame la ministre, vous n'évoquez pas les tiers, qu'il est pourtant important de masquer, me semble-t-il. En février, nous avons été très heureux de rencontrer les membres de votre cabinet, qui nous ont assuré que « que « devraient être mises en oeuvre des technologies nous assurant qu'elles pourront être déployées à brève échéance par les différents acteurs industriels auxquels le ministère envisage de recourir

Les motifs pour lesquels un préfet ou un maire peuvent instituer une interdiction de circulation ne sont aujourd'hui pas identiques. Ainsi, le préfet ne peut, en l'état du droit actuel, prévoir une telle interdiction pour des motifs liés à la qualité de l'air ou aux nécessités de la circulation. Il semblerait que cette situation pose des difficultés dans les grandes agglomérations où l'institution d'une interdiction de circulation à l'échelle de l'agglomération, sur des axes qui relèvent pour certains du pouvoir de police du préfet et pour d'autres du pouvoir de police du maire, est rendue complexe.

pouvoir, en cas de carence du maire, d'interdire ou de restreindre la circulation sur certaines voies communales pour des raisons de tranquillité publique, de protection des espèces ou des paysages. Les préfets peuvent également prendre des mesures de restriction de la circulation en cas de pics de pollution. En dehors de ces pics, je ne pense pas qu'il soit opportun de permettre au préfet de prendre des mesures d'interdiction ou de restriction de circulation sur les voies dont les maires sont gestionnaires. Cela viendrait empiéter très fortement sur les pouvoirs de police des maires dans leur commune,

Au nom du Bureau du Sénat, j'appelle chacun de vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges l'une des valeurs essentielles du Sénat : le respect, qu'il s'agisse du respect des uns et des autres ou de celui du temps de parole.

Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous dire combien nous sommes ravis de vous retrouver dans notre hémicycle ! Ma question porte sur un sujet déjà évoqué ici la hausse des frais d'inscription des étudiants extra-communautaires, qui, aujourd'hui plus encore qu'hier, suscite de grandes interrogations, voire le rejet de nombreux acteurs concernés, au premier rang desquels les présidents d'université. Cette décision, prise sans aucune concertation et dans la plus grande précipitation, n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact ; tout comme le plan Bienvenue en France, qui, certes, contient des éléments positifs, mais aurait aussi mérité d'être davantage concerté, notamment avec les collectivités territoriales. Augmenter les frais d'inscription pour les étudiants étrangers n'est pas une mesure technique. C'est un acte profondément politique, aux conséquences potentiellement lourdes pour la France et sur ce qui fait la France, parce qu'il touche aux conditions d'accès à l'enseignement supérieur, parce qu'il touche aux ressources et au financement de nos universités, parce qu'il touche, enfin, à notre diplomatie d'influence et culturelle, singulièrement à la francophonie. d'une question fondamentale, qui méritait mieux que de prendre à la hâte une telle mesure. On sait que les textes réglementaires sont prêts. Accepterez-vous de les suspendre pour prendre le temps de définir une vraie stratégie d'attractivité internationale, que vous avez voulue, monsieur le Premier ministre ?

une facilitation de l'arrivée des étudiants et un meilleur accueil, mais aussi la possibilité de soutenir le développement de formations françaises à l'international.

Le gouvernement italien a choisi de rejoindre les nouvelles routes de la soie. Toutes les routes mèneront non plus à Rome, mais à Pékin. M. Xi est ensuite allé à Monaco. Une fois n'est pas coutume, la riche principauté a accepté d'aider un État communiste. Le rocher s'apprête à accueillir la technologie 5G de Huawei, sur laquelle pèsent de lourds soupçons d'espionnage. Après l'avoir utilisée, le gouvernement américain a pris la décision d'exclure cette société. La Chine pratique un espionnage massif, y compris par le biais de ses entreprises, qui doivent, depuis une loi de 2017, contribuer au renseignement. Bien que ce pays soit le deuxième partenaire commercial de l'Union européenne, il subsiste des divergences fondamentales, notamment sur le plan des libertés individuelles ou celui du droit international. Pouvons-nous accepter que l'Empire du Milieu prenne le contrôle de la mer méridionale de Chine, au détriment de ses voisins ? Il est également regrettable que Pékin fasse pression pour empêcher Taïwan d'intégrer l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, alors que la santé est un droit humain fondamental. Nous devons être vigilants quant aux intentions chinoises, en matière de politique non seulement étrangère, mais également commerciale. La 5G chinoise ressemble à s'y méprendre au cheval de Troie : faut-il que nous lui ouvrions nos portes ? La Commission européenne doit présenter sous quinze jours une position concertée à propos de la cybersécurité des réseaux 5G. Monsieur le secrétaire d'État, quelle sera la position de la France sur ce sujet ?

Guerriau, la visite du président Xi se poursuit en ce moment même dans les murs du Sénat. C'est un moment important, un temps fort, puisque, vous le savez, nous célébrons cette année le cinquante-cinquième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays.

communes. Je constate, après un peu plus de deux jours, que cette visite a été empreinte de respect et d'amitié, sans pour autant laisser cours à la naïveté. Elle constitue une réussite pour la relation bilatérale, avec

a également rappelé les préoccupations qui sont les nôtres et celle de l'Europe sur la question des droits fondamentaux. Ce matin a d'ailleurs eu lieu un moment très important pour la rénovation du multilatéralisme, qui- vous le savez -est parfois battu en brèche par certaines puissances

pour affirmer un certain nombre d'engagements, afin que le multilatéralisme soit toujours vivace. Cela se fait dans un moment où l'Europe

La parole est à M. Laurent Duplomb, pour le groupe Les Républicains.

terminer, je vous enjoignais de ne pas faire la même erreur que Marie-Antoinette, en n'entendant pas la colère monter. Je ne pensais pas si bien dire, au vu des émeutes qui ont suivi N'oublions pas que les premières revendications de ces manifestants étaient : « Arrêtez de nous taxer ! » et « Laissez-nous vivre de notre travail ! » Par une pirouette intelligente, vous avez mis en place votre grand débat, bel écran de fumée qui, par sa durée et les interventions dithyrambiques du Président de la République, a fait oublier le coeur du sujet. Or quel n'a pas été mon étonnement en lisant les propositions du parti majoritaire et de vos ministres, prévoyant toujours plus de taxes et d'impôts augmentation des droits de succession, taxation des plus-values sur les résidences principales, retour de la taxe carbone. Aussi, monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin comprendre qu'il faut sortir de cette addiction à l'impôt ? Pouvez-vous vous engager aujourd'hui à ne créer ni augmenter aucun impôt

%. Malgré tous les prophètes de malheur, nous avons la croissance la plus élevée de l'Union européenne et nous avons terminé l'année 2018 avec une croissance de 1,6 %. Bref, tout va très bien, madame la marquise ... Il est vrai, monsieur le sénateur, que, pour baisser les impôts, il faut baisser la dépense. Or, de ce point de vue, il y a beaucoup de croyants, mais peu de pratiquants. En effet, quand nous proposons de baisser la dépense, singulièrement à la majorité sénatoriale, il y a quelques quiproquos, Je n'ai pas entendu, de la part du chef de votre parti, des propositions claires de baisse de la dépense publique, bien au contraire ! Alors, oui, notre pays doit baisser encore plus ses impôts, et c'est ce que nous faisons sur l'impôt sur les sociétés, sur la taxe d'habitation,

Madame la ministre, le 17 juillet 2017, le Président de la République fixait pour objectif le déploiement sur l'ensemble du territoire du haut débit, d'ici à 2020, ainsi que du très haut débit d'ici à 2022. Or, la semaine dernière, une enquête de l'association UFC-Que choisir estimait que 6,8 millions de Français étaient toujours privés d'un accès de qualité minimale à internet. Cela représente 10,1 % de la population. Quant au haut débit, ce sont près de 12,8 millions de Français qui en sont aujourd'hui privés, soit 19,8 % de la population. Au-delà de ces chiffres, il faut se rendre compte des importantes disparités territoriales. La même association distinguait alors deux France : celle des villes de plus de 10 000 habitants, où plus de 95 % des habitants ont accès à internet, et celle des villages de moins de 1 000 habitants, où cette proportion baisse à 69 %. à 69 %. En plus du sentiment de recul des services publics et de l'aggravation des déserts médicaux, certaines zones rurales doivent également affronter les effets d'une fracture numérique insupportable. À l'heure où la transformation numérique est le corollaire indispensable de la transformation de l'action publique, le risque est bien celui d'une désincarnation de l'administration dans ces territoires isolés numériquement. Où en sommes-nous, madame la ministre, du plan d'action en matière de couverture numérique, censé assurer une couverture en très haut débit sur l'ensemble du territoire ? Pouvez-vous nous préciser le calendrier concernant la réouverture du guichet du fonds pour la société numérique, alors que les collectivités territoriales avaient misé sur ce dispositif pour accélérer le déploiement de la fibre optique ? La parole

du réseau mobile et du réseau numérique. Le Premier ministre a d'ailleurs annoncé le déblocage de 243 millions d'euros pour huit réseaux d'initiative publique répartis sur neuf départements. S'agissant de la couverture mobile, vous connaissez l'accord que nous avons passé avec les opérateurs, sous le contrôle de l'Autorité

Le soutien de l'État aux réseaux d'initiative publique se poursuit dans le cadre du plan très haut débit, qui, je vous le rappelle, coûte 3,3 milliards d'euros

nous avons été nombreux en outre-mer à apprendre, par voie de presse, la volonté du Gouvernement de revisiter le mode opératoire des congés bonifiés, au profit des fonctionnaires ultramarins affectés dans l'hexagone. Ces congés bonifiés sont considérés comme un avantage social acquis après de dures et longues batailles. Ainsi, tous les fonctionnaires originaires des outre-mer peuvent actuellement prétendre tous les trois ans à ces congés, qui peuvent s'étaler jusqu'à soixante-cinq jours d'affilée, dont trente-cinq jours de bonification, pour rejoindre leurs familles et leurs proches. Ces congés peuvent être octroyés après trente-six mois consécutifs de service. Les fonctionnaires bénéficient en plus d'une prise en charge de leurs frais d'avion et d'une prime de vie chère tout au long de leur résidence sur leur territoire d'origine. Cette réforme devrait entrer en vigueur « à partir de 2020 », avec des congés qui seraient moins longs, mais qui pourraient être octroyés tous les deux ans au lieu de trois. De plus, une politique en faveur de la réduction du coût des billets serait mise en place. Une concertation entre les différents employeurs publics et les organisations syndicales sur cette réforme devrait avoir lieu prochainement. Il semblerait que le Gouvernement veuille aboutir, d'ici à l'été 2019, à des textes réglementaires fixant les nouvelles normes applicables en 2020 aux fonctionnaires ultramarins. Inquiète, la délégation aux outre-mer de l'Assemblée nationale a chargé David Lorion, député de la Réunion, d'un rapport sur cette réforme annoncée. En conséquence, ma question sera la suivante : pour éviter toute forme d'interprétation, pouvez-vous nous décrire en détail le contenu de cette réforme et son calendrier ?

lors de son discours en Guyane, à l'ouverture des Assises de l'outre-mer le 28 octobre 2017, le Président de la République avait annoncé une réforme des congés bonifiés. Dans le cadre de la restitution de ces mêmes assises, le 28 juin 2018, il a confirmé son intention, en annonçant une réforme du dispositif qui « sera effective sera effective à compter de 2020 pour ceux qui sont fonctionnaires, avec un principe simple : les congés seront moins longs, mais désormais tous les deux ans ». C'est avec cet objectif en tête que le Gouvernement souhaite, comme vous l'avez noté, qu'une concertation associant les organisations syndicales représentatives et les employeurs des trois versants de la fonction publique soit organisée avant l'été. Celle-ci devra permettre d'évaluer le dispositif, dont les caractéristiques actuelles ont été déterminées en 1978 et, le cas échéant, d'identifier les évolutions pertinentes. En toute hypothèse, et j'insiste sur ce point, conformément aux annonces du Président de la République, les travaux seront conduits non pas pour remettre en cause le droit au congé bonifié, mais pour en moderniser les modalités d'application, de façon à permettre aux personnes concernées de bénéficier de congés plus fréquents, tout en répondant aux enjeux d'efficacité et de continuité des services publics. Le régime actuel des congés bonifiés n'est en réalité plus adapté, ni à notre temps, ni à nos modes de transport, ni même à nos modes de congés, et il mérite d'être revu. Nous souhaitons une politique qui incite à revenir plus vite, plus facilement, plus souvent et moins longtemps, comme l'a annoncé le Président de la République. Ainsi, nous souhaitons que, au lieu de partir tous les trois ans, comme c'est le cas aujourd'hui et vous l'avez rappelé, les agents publics de l'hexagone qui ont leurs intérêts matériels et moraux dans les territoires d'outre-mer puissent partir tous les deux ans, avec leur famille, et ce dès l'année 2020. Pour celles et ceux qui ont bénéficié de ce système en 2018, cela permettra de démontrer la rapidité de la nouvelle rotation.

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale, et j'y associe mon collègue Gérard Longuet. Elle porte sur la place réservée à la bataille de Verdun dans les nouveaux programmes scolaires, à la suite du débat passionné de ces derniers jours.

Monsieur le ministre, si vous avez réaffirmé que la bataille de Verdun continuerait bien à être étudiée en cours d'histoire par les élèves de première, nous souhaitons qu'elle soit plus explicitement nommée dans le, au même titre que la bataille de la Somme. Verdun est un symbole de la Grande Guerre, un haut lieu d'histoire où tant d'hommes se sont sacrifiés. Les nouvelles générations viennent en nombre sur ce site chaque année. Le champ de bataille de Verdun porte encore les stigmates de l'horreur. Cette zone rouge d'environ 15 000 hectares au paysage défiguré, où reposent encore près de 100 000 soldats, et les vestiges de neuf villages détruits reconnus « morts pour la France », témoigne de l'enfer de Verdun. Verdun est aujourd'hui devenu la capitale mondiale de la paix et le symbole de l'amitié franco-allemande. En attestent la poignée de main historique entre Helmut Kohl et François Mitterrand la visite d'Angela Merkel et de François Hollande en 2016. Au lendemain de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre et à quelques semaines des élections européennes, il me semblait nécessaire de le souligner. Verdun porte de le souligner. Verdun porte un message d'universalité contemporain, qui doit absolument être transmis à notre jeunesse. Si nous pouvons faire confiance à l'appréciation de nos professeurs, pouvez-vous malgré tout nous rassurer quant à son inscription officielle dans les programmes scolaires ?

La Première Guerre mondiale elle-même n'était pas réellement décrite, puisqu'elle était là simplement à titre d'exemple de ce qu'était une guerre totale absolue. Les nouveaux programmes sont incontestablement un progrès à cet égard et à bien d'autres, puisqu'ils sont chronologiques. On étudie la Première Guerre mondiale de façon chronologique,

Selon moi, Verdun n'est pas morte ! Il y a eu une première victoire, et, si la mémoire est une victoire, alors il y aura justement une seconde victoire de Verdun.

À l'évidence, en matière de déclaration et de promesse gouvernementale, le principe de précaution s'impose : comme le dit le bon sens populaire, « quand c'est flou, il y a un loup Dernière annonce en date, l'assouplissement des règles de cumul emploi-retraite, permettant aux retraités de continuer de travailler, afin d'obtenir des points supplémentaires pour leur trop faible pension. C'est aberrant, dans un contexte de chômage de masse et de révolution numérique, qui appelle une réduction du temps de travail, et d'une espérance de vie en bonne santé bien au-dessous de la moyenne européenne. En effet, il va falloir travailler plus longtemps, car le système de retraite par points que vous voulez mettre en place conduira à une baisse des pensions de retraite, qui affectera particulièrement les ouvriers et les femmes. Dans ces conditions, il faudra donc bien travailler plus pour s'assurer des revenus décents. Vous continuez les annonces dans le plus grand flou et vous faites fi des concertations en cours avec les partenaires sociaux, mais une chose est sûre : les Français en ont assez de voir leurs droits attaqués sous des prétextes financiers. C'est d'ailleurs ce que révèle un sondage récent de l'institut Harris, selon lequel presque deux tiers de nos concitoyens sont opposés à un allongement de la durée de cotisation et au report de l'âge légal de départ à la retraite. Nous savons ce que pensent les Français. Peut-on enfin savoir comment se positionne le Gouvernement et quelles sont ses réelles ambitions concernant les retraites ? Très

démographique majeur, comme il y en a peu dans l'histoire des sociétés. Le vieillissement de la population représente un défi majeur pour notre protection sociale et pour son financement, notamment pour notre système de santé et de prise en charge des personnes âgées dépendantes. Il nous faudra déployer des moyens financiers considérables

mais pouvez-vous affirmer que les travailleurs pourront toujours partir à taux plein à soixante-deux ans, alors que tout montre que votre objectif inavoué est bien le recul de l'âge de départ en retraite ?

Vous avez récemment déclaré, dans le journal, que vous vous battrez pour chaque emploi industriel menacé. Quelle belle déclaration ! Or vous voilà confronté, dans la Sarthe, à des travaux pratiques ; c'est le moment de passer des intentions aux actes.

Vu la situation actuelle, le moins que l'on puisse dire est qu'il a singulièrement manqué de clairvoyance ... À situation exceptionnelle, nous attendons un traitement exceptionnel. La présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morançais, est prête à engager sa collectivité pour contribuer au sauvetage de cette industrie et des emplois qui y sont attachés. Quelles initiatives comptez-vous mettre en oeuvre, de manière urgente, pour accompagner la région, et pour que votre priorité affichée- sauver les emplois industriels -soit une réalité dans la Sarthe ? Comment entendez-vous prendre en compte le caractère exceptionnel du dossier Arjowiggins ?

à la suite du placement en redressement judiciaire de ces trois sites. C'est grâce à l'État que l'exploitation a pu se poursuivre ; c'est également grâce à lui que plusieurs repreneurs ont présenté un dossier sur les sites de Château-Thierry et du Bourray. En outre, vous le savez, un repreneur avait présenté un dossier concernant les trois sites. Mercredi dernier, ce repreneur a indiqué qu'il n'était pas en mesure de rassembler l'ensemble des

l'argent public est aujourd'hui réuni pour faire face à cette reprise. Nous sommes aux côtés des salariés et des organisations syndicales pour trouver une solution ; il reste 20 millions d'euros, d'origine privée, à trouver. Or, cela, c'est beaucoup plus difficile, et cet argent ne pourra pas faire l'objet d'une garantie de l'État- ce sont les règles du jeu.

plus en plus d'agriculteurs adoptent ce mode de production, qui répond aux attentes de nos concitoyens et qui contribue à la préservation de la santé humaine, de l'environnement, de la biodiversité, mais aussi

Tout comme les acteurs historiques de cette filière, je me réjouis de cette prise de position, qui ne me surprend pas, mais j'attends de savoir si ces déclarations seront suivies d'actes politiques forts et immédiats. Le 3 avril prochain, votre gouvernement sera appelé à se prononcer, au sein du Comité national de l'agriculture biologique, sur la question de la production en bio de fruits et légumes sous serres chauffées. L'enjeu de cet arbitrage est d'interdire le label bio aux légumes produits à contre-saison, tels que les tomates en hiver. Les autres États européens encadrent encore peu ces pratiques ; c'est donc à la France d'envoyer un signal fort, en montrant l'exemple et en défendant cet encadrement auprès de l'Union européenne. Cet arbitrage,

pour la production à contre-saison de légumes labellisés bio ? La parole

: à la surtransposition et au fait de nous mettre en difficulté économique par rapport à d'autres pays. La France est un pays leader dans l'agriculture biologique, nous devons continuer à l'assumer. Évidemment, cultiver des légumes et des fruits hors saison ne correspond pas à ce que nous devons faire dans le cadre de l'agroécologie- c'est pourquoi j'ai indiqué que je n'étais pas favorable à l'agriculture industrielle biologique, et c'est la position du Gouvernement

appelée « Hauts-de-France propres », a connu un réel succès, rassemblant 50 000 de nos concitoyens sur toute la région. Cette manifestation volontaire, solidaire et écologique a malheureusement été entachée par une pollution d'origine maritime, survenue quelques jours auparavant, sur le littoral du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.

Cela est dû- nous le savons tous -au nettoyage de cuves de chimiquiers. Madame la secrétaire d'État, la semaine dernière, le Gouvernement fut interpellé au sujet du. À cette occasion, il fut déclaré que des propositions seraient faites à l'échelon européen pour renforcer la sécurité et la réglementation. Il y a urgence ! Quels recours techniques et judiciaires comptez-vous engager afin de pénaliser les contrevenants au maintien de la biodiversité de l'un des détroits les plus fréquentés du monde et de notre littoral ?

Effectivement, nous avons été alertés le lundi 18 mars dernier sur l'existence de dizaines de boulettes de paraffine sur les côtes, depuis Fort-Mahon, dans la Somme, jusqu'à Marck-en-Calaisis, dans le Pas-de-Calais. Des associations se sont mobilisées dès le week-end des 16 et 17 mars, afin de nettoyer les plages. Je veux d'ailleurs saluer la mobilisation des associations, des communes et des citoyens ; environ 200 litres de paraffine ont pu être récupérés dans cette opération de nettoyage. entendu immédiatement mobilisé ; les directions départementales des territoires et de la mer de la Somme et du Pas-de-Calais ont effectué des prélèvements et mené des analyses toxicologiques sur ces prélèvements. Ces analyses sont rassurantes

à quatorze heures, les habitants du quartier de la Bricarde ont été pris en otage sous les feux croisés de kalachnikov d'un commando d'une dizaine d'hommes encagoulés et portant des brassards de police, sortis de trois véhicules, dont certains étaient dotés de gyrophare. Alertée par des mères hurlant de peur face à ces scènes de guerre, j'ai été saisie d'un mélange de colère et d'indignation. Trois quarts d'heure, c'est le temps qu'il a fallu aux forces de l'ordre pour arriver sur place. Pendant ce temps, les habitants, dont des enfants, essayaient d'échapper aux balles de ces armes de guerre.

L'approche globale, mise en place en 2012 et conduite par vous-même, monsieur Nunez, a porté ses fruits, mais elle a été abandonnée, laissant place à la recrudescence des trafics et à la violence qui les accompagnent.

Ma question s'adressait à Mme le ministre des solidarités et de la santé. Lorsqu'Emmanuel Macron était candidat à la présidence de la République française, il ne cessait de souligner l'impérieuse nécessité de faire montre d'une transparence totale quant aux affaires publiques. Pourtant, cette déclaration d'intention n'est pas toujours suivie d'effet lorsqu'une question est susceptible de mettre le Gouvernement en difficulté. Ainsi, la semaine dernière, dans cet hémicycle, le secrétaire d'État Adrien Taquet a refusé de répondre clairement lorsqu'il fut interpellé par notre collègue Nathalie Goulet au sujet de la fraude massive sur les cartes Vitale.

Nous sommes en droit de connaître le nombre total de ces numéros et le nombre de ceux qui sont encore actifs. Je souhaite aussi que vous nous précisiez le nombre de numéros d'inscription au répertoire qui ont été attribués à des étrangers résidant en France. En effet, l'opacité singulière que vous persistez à entretenir sciemment nous interpelle. Si j'attends une réponse précise, je désire surtout que vous m'indiquiez les mesures que vous envisagez de prendre afin de remédier à la fraude massive sur les utilisations de la carte Vitale. La parole

à cause d'un numéro de sécurité sociale, le NIR, attribué sur le fondement de faux documents à des assurés sociaux nés hors de France. Ces chiffres sont souvent relayés, et l'on comprend l'inquiétude qu'ils peuvent susciter, tant le préjudice subi serait important. La ministre Agnès Buzyn a rapidement demandé que ces données soient examinées. Au regard des compléments qui ont été apportés, je puis vous affirmer que ces chiffres ne correspondent en rien à la réalité. Il me semble par conséquent nécessaire de rétablir les faits. Il serait en effet regrettable que de fausses informations amènent certains de nos concitoyens à stigmatiser les personnes nées à l'étranger, en les associant à des fraudeurs, ou à imaginer que les prestations de sécurité sociale sont versées sans aucun contrôle, donc sujettes à un phénomène massif de fraude.

qui visait à évaluer la conformité des pièces justificatives acceptées par le service administratif national d'immatriculation des assurés au cours du processus d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire. Il ne s'agit donc pas de fraudes avérées, puisque les assurés dont les pièces présentaient des anomalies ont été recontactés et ont pu apporter des pièces justificatives justificatives complémentaires. Dans la plupart des cas, il n'y avait pas d'intention de fraude chez ces assurés. Une mission d'évaluation et de contrôle sur la fraude à l'obtention de numéros de sécurité sociale, présidée par le rapporteur général, est en cours depuis deux mois ; elle devrait rendre ses premières conclusions au cours des semaines qui viennent.

Une fois encore, votre refus de répondre clairement à une question simple résonne comme une caution apportée aux fraudeurs, d'autant que leurs méfaits portent sur des sommes considérables. Nos compatriotes, sur lesquels vous avez accru la pression fiscale, apprécieront certainement.

pour ce qui concerne la régulation des plateformes d'intermédiation numérique entre clients détenteurs de fret et entreprises de transport routier de marchandises. Ces plateformes mettent en relation des clients qui possèdent des colis à transporter et des entreprises de transport ou des travailleurs

entre les actuels commissionnaires de transport et les plateformes numériques, qui agissent dans le même champ, mais ne sont pas soumises à la même réglementation. Il est ainsi proposé de considérer les plateformes numériques officiant en tant qu'opérateurs de transport de marchandises comme des commissionnaires de transport. Autrement dit, puisque les activités exercées par les plateformes numériques de fret sont en tout point similaires à celles des commissionnaires de transport, cet amendement vise à leur appliquer ce statut.

entre clients détenteurs de fret et entreprises de transport public routier de marchandises. Pour nous assurer que le transport motorisé n'est pas le seul concerné, nous souhaitons inclure dans le champ de cette ordonnance les livreurs professionnels effectuant des déplacements à vélo ou à pied.

le champ d'application de l'ordonnance, afin qu'elle concerne les transporteurs routiers de personnes lorsqu'ils effectuent du transport de marchandises à titre accessoire. En effet, cette activité se développe de plus en plus. Ainsi, des cars transportant des personnes profitent de la place libre dans leur coffre pour transporter des marchandises. Il s'agit d'encadrer une telle activité.

est l'avis de la commission ? Il est nécessaire d'encadrer l'activité des plateformes d'intermédiation numérique spécialisées dans le transport de marchandises, qui agissent aujourd'hui sans cadre juridique clair- c'est une évidence -, afin notamment de définir leurs responsabilités en fonction de leur niveau d'intervention dans la relation commerciale, entre les clients détenteurs de fret et les entreprises de transport.

vise à soumettre l'ensemble des plateformes d'intermédiation numérique spécialisées dans le transport de marchandises au statut de commissionnaire de transport, ce qui ne permettrait pas de prendre en compte la diversité de leurs natures et de leurs activités. En effet, certaines plateformes interviennent directement dans la relation commerciale entre le client détenteur de fret et l'entreprise de transport, en définissant, par exemple, les conditions d'exécution de la prestation de transport et sa tarification. Leur activité s'apparente donc à celle d'un commissionnaire de transport, tandis que d'autres plateformes se contentent de mettre en relation les clients et les entreprises de transport sans intervenir dans la relation commerciale. Tel est le cas des bourses de fret numérique. Ainsi, leur appliquer le statut de commissionnaire de transport ne serait pas approprié.

qui prévoit que l'ordonnance porte sur les conditions d'exercice de l'activité des plateformes d'intermédiation numérique spécialisées dans le domaine du transport de marchandises, ce qui englobe les livraisons de marchandises à vélo ou à pied, ainsi que la livraison au moyen de véhicules qui ne sont pas des véhicules de transport de marchandises.

est non pas de mettre en relation un donneur d'ordres et un transporteur, mais de trouver, pour le compte d'un donneur d'ordre, avec des moyens qu'il lui appartient de trouver,

des plateformes d'intermédiation pour le transport de marchandises. Face au risque de concentration de ces plateformes, cette régulation sur les modalités d'échanges et les tarifs des prestations se doit d'être négociée dans le cadre d'une convention collective de branche. Afin de garantir l'aboutissement effectif de ces mesures de régulation, une mesure supplémentaire supplétive est prévue en cas d'échec de la négociation dans le délai prévu par la loi. Quel par la loi. Quel est l'avis de la commission ? Renvoyer à un accord de branche du secteur routier le soin de définir les conditions d'exercice des plateformes d'intermédiation numérique, dont l'activité ne relève pas aujourd'hui du secteur du transport routier,

de cyclomoteurs et de cycles à pédalage assisté, afin qu'ils relèvent d'une législation différente de celle applicable aux conducteurs d'utilitaires de 3,5 tonnes. Cela peut paraître logique au regard de la différence des véhicules. Aujourd'hui, pourtant, les conditions d'accès à la profession de transporteur routier de marchandises sont trop complexes pour ceux qui utilisent des scooters et des vélos électriques. Ces obstacles poussent d'ailleurs certains livreurs à contourner les règles existantes et à s'inscrire sur les plateformes de livraison en déclarant un vélo, alors qu'en réalité ils utilisent un scooter. Ils ne sont donc pas assurés et le moindre accident peut se terminer en drame. Il convient de les protéger et d'encadrer ces nouveaux usages. J'ajoute que la plupart d'entre eux sont jeunes et n'ont pas toujours les ressources financières nécessaires pour obtenir la capacité professionnelle. Dans les conditions actuelles, on les prive donc de travail. C'est pourquoi il convient d'assouplir les conditions d'accès à la profession de transporteur public pour ces deux types de véhicules. Le développement des deux-roues et des vélos cargo à assistance électrique est une occasion à saisir pour relever le défi des nouvelles mobilités,

du transport de marchandises. En revanche, l'activité de transport de marchandises par cyclomoteurs est soumise à ce statut et aux obligations qui en découlent. S'ils étaient adoptés, ces amendements excluraient de la réglementation applicable aux transporteurs routiers toutes les entreprises utilisant de tels véhicules.

de toute obligation d'inscription au registre des entreprises de transport, ce qui déstabiliserait totalement le marché du transport routier et serait au demeurant en contradiction avec la réglementation européenne. avec la réglementation européenne. Les entreprises qui utilisent uniquement des cycles à pédalage assisté ne sont pas soumises à l'obligation d'inscription au registre des entreprises de transport. En revanche, les cyclomoteurs le sont, ce qui renvoie à un objectif de professionnalisation du secteur de la course. Selon moi, il n'est pas opportun de dispenser les entreprises utilisant des cyclomoteurs de répondre à des exigences d'honorabilité,

est à Mme Catherine Dumas, sur l'article. L'article 18 renforce la régulation des opérateurs qui mettent à disposition des utilisateurs des engins ou véhicules accessibles en libre-service et sans station d'attache, suivant le système de. J'ai souhaité intervenir en introduction de notre discussion sur cet article, car j'ai le sentiment qu'un certain nombre d'amendements qui vont être défendus et dont nous débattrons trouvent leur origine et, sans doute, leur solution dans le fait que les engins de mobilité qui font l'objet de notre attention n'ont pas de station d'attache.

Toutes ces préoccupations, et d'autres encore, comme l'organisation de l'espace public, seraient apaisées si les engins restaient accessibles en libre-service, mais avaient une station d'attache. plus oublier la nécessaire recharge énergétique des appareils : comme elle ne peut s'effectuer que sur base, elle doit être organisée l'enlèvement et la repose nocturnes des véhicules

Il convient de la réguler, afin de profiter des effets bénéfiques liés aux nouveaux services de mobilité tout en limitant les effets néfastes pour l'ordre public et la sécurité de tous. Des règles sont nécessaires pour permettre un développement harmonieux et sain des nouvelles mobilités décarbonées, mais ces règles ne doivent pas venir freiner le développement de ces nouvelles offres, plébiscitées par les usagers.

Cela va sans doute freiner l'innovation et empêcher de nouveaux acteurs de se développer, en cas de décision arbitraire de la ville, ou d'évoluer, en cas d'exigences trop strictes. Cela soulève également un problème de concurrence déloyale, dans le cas où les pouvoirs publics locaux offriraient leurs propres services de.

Dans la majorité des cas, les opérateurs préviennent les communes de leur implantation. Ils sensibilisent les usagers aux enjeux de la sécurité routière, par le biais des applications. Certains distribuent même des casques gratuitement. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous vous proposerons de revenir à la rédaction initiale de cet article, qui laissait une plus grande marge de manoeuvre aux AOM et un contrôle de ces acteurs. Permettre aux AOM de réguler ces derniers à l'échelle de chaque territoire garantira, sans doute, une meilleure régulation, ainsi qu'un contrôle plus efficace. La sensibilisation à la sécurité, concernant l'usage de ces nouveaux services, n'en sera que plus efficace. Mes chers collègues, l'enjeu est de taille : ne nous laissons donc pas piéger par l'impatience et la volonté d'aller trop vite ! Ces nouvelles mobilités sont sans doute l'avenir ; elles doivent permettre à chacun de se déplacer librement, notamment pour effectuer le dernier kilomètre.

Le texte adopté par votre commission introduit un régime d'autorisation préalable pour les opérateurs de services dits « de », adossé à la mise en place d'une redevance d'occupation temporaire du domaine public par engins ou par véhicules.

Par ailleurs, je suis convaincue que le rôle des collectivités propriétaires du domaine public est essentiel dans le dispositif. Néanmoins, je voudrais souligner plusieurs difficultés. Je ne pense pas, d'une part, que l'instauration systématique d'un régime d'autorisation préalable soit adaptée. Certaines collectivités pourraient simplement souhaiter définir un ensemble de règles, ou un cahier des charges à respecter, sans avoir à suivre une procédure administrative d'autorisation, voire de sélection, ce qui est la règle de droit commun dès lors qu'il y a autorisation d'occupation du domaine public. Je suis, d'autre part, convaincue que l'autorité organisatrice doit jouer un rôle plus central dans le dispositif, notamment pour les services qui n'utilisent pas le domaine public au-delà des places de stationnement déjà disponibles. Nous poursuivrons la concertation en tenant compte des orientations du Sénat, afin de construire un dispositif qui donne toutes leurs places aux autorités organisatrices comme aux communes, chacune dans leur champ de compétence, qui offre de la souplesse, de manière à éviter des procédures administratives coûteuses tant pour les acteurs économiques que pour les administrations, et qui facilite le développement de nouveaux services, tout en tenant compte des problématiques de sécurité, de stationnement et d'aménagement urbain, et en évitant la fragmentation des règles. En attendant le résultat de ce travail, qui est engagé et qui se poursuit avec les différents acteurs, le Gouvernement propose, au travers de cet amendement,

possibilité de mettre en place un régime d'autorisation préalable pour les opérateurs de, notamment par le biais d'une liste de prescriptions relatives aux caractéristiques des engins et aux mesures prises en matière de règles de circulation ou de retrait des véhicules défaillants. cet amendement, nous proposons d'aller plus loin que le système d'autorisation préalable et de mettre en place un dispositif de délivrance de licences d'exploitation pour les plateformes de véhicules en partage. Cette licence serait délivrée par les EPCI et les communes ; elle couvrirait tout ou partie de leur ressort territorial, et serait soumise à un renouvellement annuel sur demande de l'opérateur. Du fait du caractère fortement concurrentiel de ce marché et de son évolution rapide, il est en effet pertinent d'instaurer une forme de clause de revoyure, afin d'inciter les collectivités à examiner régulièrement sur cette question et à sélectionner les opérateurs les plus pertinents en la matière. L'amendement

que les opérateurs des nouveaux services de mobilité devront respecter sous peine de sanctions. Elles pourront s'emparer du sujet, si elles le souhaitent, sans freiner le développement des opérateurs et des nouveaux services de mobilité. Tel est le sens de cet amendement. L'amendement n° 317 rectifié,

À cette fin, y figure une série de prescriptions exclusives dont ne peuvent se départir les autorités compétentes, alors même que cette liste pourrait se révéler inadaptée sur certains territoires, en raison de spécificités locales. Le présent amendement tend donc à laisser le soin aux collectivités de définir quelles prescriptions elles souhaitent édicter, afin d'adapter au mieux l'offre proposée aux besoins en mobilité de la population, tout en respectant le partage équitable et harmonieux de l'espace public, sans oublier les plus fragiles, et en évitant d'offrir une image d'anarchie et de ville mal tenue. La parole

sur l'article. Cet article réglemente l'activité des cycles à pédalage assisté assurant le transport de personnes. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a renforcé le dispositif de régulation des vélos-taxis en les soumettant à un régime d'autorisation préalable, mais aussi à des conditions d'honorabilité professionnelle et d'aptitude à la conduite des conducteurs. Les modifications apportées par la majorité sénatoriale vont dans le bon sens. Pour autant, dans sa nouvelle rédaction, n'apporte pas de garanties suffisantes aux conducteurs des vélos-taxis, dont le nombre est estimé à quatre cents dans la capitale et dont la dureté du travail n'est ni reconnue ni prise en considération, entraînant un risque d'exposition à l'épuisement professionnel, mais également des dangers pour la santé, à cause de l'absorption en grande quantité de particules fines, puisqu'ils se trouvent au même niveau que les pots d'échappement des véhicules motorisés. En matière de sécurité, le port du casque devrait être obligatoire pour le conducteur comme pour les passagers, afin de réduire les conséquences des accidents de la route. À partir du moment où les conducteurs utilisent leur cyclomoteur pour un usage exclusivement commercial, une plaque d'immatriculation devrait être obligatoire, tout comme la souscription d'une assurance de type cyclomoteur et la détention du code de la route. Bref, les conditions de sécurité sont loin

étant donné la faible puissance de ces engins. Nous avons voulu encadrer et moraliser- j'ose le mot -cette pratique. Étendre ce régime simplifié aux cyclomoteurs, dont la puissance est supérieure et qui présentent donc davantage de risques pour les usagers, ne me paraît pas opportun. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable

en tant que véhicules motorisés à deux ou trois roues. Je ne pense pas qu'il soit souhaitable d'alléger cet encadrement non plus que de permettre aux véhicules

en particulier celles du droit du social. « L'intermédiation numérique » comme activité spécifique justifierait une telle mise à l'écart : il y aurait non plus des « travailleurs », encore moins des « salariés mais des « utilisateurs » ou des « prestataires extérieurs » ; non plus des « employeurs », mais des « intermédiaires » ; non plus des sanctions directes, mais des incitations. Et la désactivation fait figure de rupture contractuelle euphémisée. Il ne s'agit pourtant que d'une torsion de la réalité opérée par le recours à un langage spécifique. Dans les faits se multiplient les pratiques de concurrence déloyale envers les entreprises qui respectent la loi et une vaste opération de dumping social La Cour de justice de l'Union européenne est pourtant formelle : l'intermédiation numérique n'est que la modalité d'exécution d'un service qui dépasse la simple mise en relation. Si Uber est une société de transport, Deliveroo une société de livraison de repas, ces plateformes ont besoin des travailleuses et des travailleurs qui réaliseront, pour leur compte, l'activité économique et commerciale qu'elles encadrent et dirigent. C'est ce que l'on appelle du travail salarié. Or le développement des plateformes numériques de travail est l'occasion d'une paupérisation terrible des travailleuses et des travailleurs, qui restent à l'écart du statut de l'emploi et sont payés à la tâche, sans assurance maternité, chômage, vieillesse ou maladie, sans protection contre le pouvoir de contrôle, de direction et de sanction des plateformes, et soumis à la loi du plus fort. Pour protéger ces travailleurs, lutter contre le faux travail indépendant, le dumping social et les pratiques de concurrence déloyale, il semble indispensable d'établir bien plus qu'une charge,

! Ce n'est donc pas avec une charte facultative, même bien pensée, que l'on réglera ces questions. Si elle était adoptée dans le domaine des transports, il est évident qu'elle ferait jurisprudence

Les fortes perspectives de développement du secteur et la fréquence des conflits sociaux en son sein appellent une réaction. Mes chers collègues, il incombe aux responsables politiques de prendre acte des changements profonds qu'opère la révolution numérique au sein de notre société et de les accompagner. La sécurisation de la relation entre les plateformes et les travailleurs indépendants et le développement de la responsabilité de ces plateformes doivent être une priorité.

Les effets bénéfiques de cet article sont nombreux, le rapporteur l'avait lui-même reconnu lors de l'examen en commission : de meilleures conditions d'exercice de l'activité des travailleurs, des garanties de protection sociale, la sécurisation des parcours professionnels. Cet article répond donc à un double enjeu : le besoin de sécurisation des relations entre les plateformes et les travailleurs, d'une part, le besoin de moralisation du secteur par le renforcement des garanties sociales offertes à ces travailleurs, d'autre part. Vous l'aurez compris, ces dispositions doivent être un vecteur de sécurité juridique, tout en encourageant les plateformes à adopter de bonnes pratiques dans leurs relations avec leurs salariés. Il convient de continuer les travaux sur cette question et de légiférer de façon posée. Je pense que l'enjeu auquel nous faisons face est moins de trouver des moyens de requalification en salariat que d'imaginer des protections adaptées à ces nouvelles formes de travail, qui correspondent à des évolutions profondes de notre société.

Par conséquent, nous ne devons pas entraver leur développement. Bien plus, nous devons le faciliter. Pour autant, il n'est pas acceptable que, au prétexte qu'ils sont indépendants, les travailleurs des plateformes soient dépourvus de protection et de droits.

qui souhaitent organiser librement leur travail, et aux attentes des plateformes, qui, pour fonctionner, doivent pouvoir correctement fixer certaines obligations. À ce titre, l'article 20, tel qu'il vous est présenté, constitue une première étape.

notamment dans le domaine des transports où des règles de sécurité doivent s'appliquer, comment répondre aux aspirations des chauffeurs en termes de rémunération, comment encadrer davantage les conditions d'exercice des plateformes et leur ouverture de données ? Il s'agit là d'un premier pas.

reprend l'article 66 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, introduit en séance publique par le rapporteur de l'Assemblée nationale, puis censuré par le Conseil constitutionnel, qui l'a considéré comme un cavalier législatif.

nous considérons qu'une telle charte, qui, rappelons-le, ne serait que facultative, est évidemment largement insuffisante pour garantir pleinement les droits des travailleurs ultraprécaires qui sont surexploités par ces plateformes. vous venez de nous peindre un paysage idyllique, dans lequel des jeunes rêveraient de ne plus être salariés et de recourir au travail ces plateformes.

à la décision de la Cour de cassation, qui, au mois de novembre 2018, a estimé que les livreurs à vélo de Take Eat Easy devaient être salariés, car ils sont dans un lien de subordination par rapport à la plateforme, ou, plus récemment à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 janvier 2019, qui a requalifié le contrat liant un ancien chauffeur VTC à la société Uber en contrat de travail, jugeant là aussi qu'il existait un faisceau d'indices suffisant caractérisant le lien de subordination et renvoyant donc l'affaire devant le conseil des prud'hommes. Si nous adoptions cet article en l'état aujourd'hui, nous empêcherions ces salariés de faire entendre justice, comme les deux exemples que je viens de citer. Nous proposons donc la suppression de cet article. La seule façon de reconnaître les droits de ces travailleurs, c'est évidemment le salariat qui n'a absolument rien

Il ne semble pas opportun de légiférer sur un dispositif facultatif qui, en l'état, semble avant tout sécuriser les plateformes. De surcroît, le contenu des chartes sera rédigé par ces dernières, qui sauront utiliser, le cas échéant, les subtilités rédactionnelles au détriment des chauffeurs. Au surplus, les plateformes s'appuient déjà sur un règlement intérieur que les chauffeurs doivent accepter et respecter. Dès lors, il est préférable de ne pas alourdir inutilement le texte avec un dispositif

qui soit concédé en la matière. En effet, face aux risques attestés de requalification des prestations des travailleurs indépendants de ces plateformes en salariat, comme c'est le cas actuellement devant différents tribunaux, en France et à l'étranger, du fait du lien de subordination qui lie les livreurs ou les VTC à ces plateformes de mise en relation avec leurs clients, cette mesure non contraignante de sécurisation est tout à fait relative juridiquement, puisqu'un travailleur indépendant peut toujours tenter une action individuelle devant les prud'hommes.

que c'est un premier pas, nous ne sommes pas prêts à le franchir. Les plateformes ont détourné le statut d'autoentrepreneur pour échapper au salariat. Or ce qui détermine le salariat, ce sont les conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie, et, même si, selon vous, madame

cet article n'est ni suffisant ni de nature à régler la véritable difficulté que posent la jurisprudence récente de la Cour de cassation ou l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en requalifiant en contrat de travail la relation qui lie les

visant à définir un statut spécifique et des droits spécifiques pour ces travailleurs, afin de sortir du flou juridique insécurisant pour tous les acteurs, y compris les clients. C'est d'ailleurs ce que montrent les amendements de repli n 619 rectifié ,

S'il faut prendre acte du fait que certains travailleurs de ces plateformes ont souhaité une requalification, je puis vous assurer que je passe un certain temps avec ces travailleurs, notamment dans le domaine des VTC ou dans d'autres domaines, et que, de façon

ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas un statut de salarié qu'il faut les priver des droits prévus à l'article 20, notamment en termes de formation. Il nous faut inventer des droits pour des travailleurs de plateformes qui ne veulent pas être des salariés.

souplesse, de la diversité des situations, de leur caractère non récurrent et imprévisible, demandent une adaptation du travailleur au service du client.

la demande, et la souplesse de l'autoentrepreneur ou du travailleur indépendant, qui accepte, lui, pour des raisons qui lui sont propres, des contraintes qui ne sont en général pas imaginées pour des activités à statut,

de la majorité sénatoriale de bien réfléchir à cette évidence : il faut choisir le travail ... L'exploitation

cette logique du moins-disant. Je lui ai expliqué ce que pourrait lui apporter un nouveau statut, telle une coopérative d'activités et d'emplois. Je le répète : on peut être entrepreneur salarié à temps partiel, en CDI, et peser collectivement face aux plateformes. Sinon, on est atomisé, explosé, ubérisé, puis, un jour, déconnecté. Le problème de fond de certaines plateformes est que leur modèle économique ne permet pas une juste rémunération du travail.

présenté par le Gouvernement dès le début du quinquennat. L'exposé des motifs du présent projet de loi fait état des ambitions du Gouvernement. Néanmoins, pour leur donner toute leur force et les traduire par une action résolue

De nombreux pays s'engagent eux aussi à mettre fin à la commercialisation des véhicules qui roulent à l'essence et au diesel : le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, l'Irlande et l'Inde en 2030, le Royaume-Uni et l'Espagne en 2040. En les rejoignant, la France, troisième producteur automobile en Europe, pèsera de tout son poids sur le continent, pour sortir des énergies fossiles et accélérer la transition du secteur automobile, pilier de l'économie européenne. À quelques semaines des élections européennes, ce signal fort permettra non seulement d'assurer une visibilité à long terme aux acteurs de la filière, d'accompagner les évolutions liées à cette transformation inéluctable et ses impacts sur l'emploi, mais également de répondre aux problématiques de la pollution de l'air et de ses conséquences sanitaires très importantes.

vise à inscrire clairement dans la loi l'interdiction de la vente des véhicules thermiques à l'horizon de 2040. Cette inscription est parfaitement cohérente avec l'objet de ce projet de loi, qui privilégie les mobilités alternatives. Elle est indispensable alors que la prochaine loi générale sur l'organisation des transports risque de se faire attendre vingt ou trente ans. Cette mesure est demandée par toutes les ONG environnementales et par nombre de nos concitoyens, qui se sont exprimés lors du grand débat ou qui participent chaque semaine, chaque mois aux marches pour le climat. Il faut en finir avec les véhicules thermiques pour les deux raisons fondamentales que nous avons déjà évoquées à plusieurs reprises. L'Irlande, la Suède, les Pays-Bas et le Danemark l'ont déjà fait fait ; la France doit embrayer et montrer l'exemple. C'est rendre service à nos constructeurs que de leur fixer un cap clair. C'est favoriser l'innovation et s'assurer que nos fleurons industriels, pleinement tournés vers l'avenir, auront un temps d'avance sur la concurrence.

Nous savons que la France s'est fixé des objectifs ambitieux, afin de réduire la place de la voiture thermique. Il convient maintenant de passer des prises de position aux actes en fixant dans la loi une date ferme de fin des ventes de nouveaux véhicules thermiques, l'année 2040. Cette inscription apparaît comme l'un des moyens d'inciter l'ensemble de la filière automobile à progresser encore plus rapidement dans la recherche de solutions de

Le présent projet de loi est réellement l'occasion d'envoyer un message fort, en particulier si nous voulons limiter le réchauffement à 1,5° et répondre avec responsabilité au message que nous envoient à nous, responsables politiques, les marcheurs pour le climat, en particulier les jeunes générations.

dans la loi l'objectif de la fin de la vente des véhicules neufs diesel et essence à l'horizon de 2040. En effet, il est temps de prendre des engagements forts : n'est-ce pas la philosophie même de cette loi ? Franchissons le pas Il s'agit de favoriser le remplacement progressif de la flotte de véhicules diesel et essence par des véhicules à faibles émissions, car le but, ne l'oublions pas, est de répondre aux problématiques de pollutions de l'air et de leurs dramatiques conséquences tant sanitaires qu'environnementales. Il est nécessaire d'être dans la clarté une vision de l'avenir proche pour enclencher la transformation de la société propre à remédier à ces problèmes, dont, à lui seul, le réchauffement climatique est le plus emblématique. En France, le nombre d'immatriculations de véhicules électriques, s'il a augmenté, reste dérisoire par rapport au nombre total d'immatriculations. Si l'on se réfère à la part des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans le total des ventes 2018, les 2,1 % de la France font pâle figure, loin derrière nos partenaires européens comme la Norvège, la Suède, les Pays-Bas, le Portugal. Je me permets de rappeler que la Norvège s'est fixé comme objectif d'interdire la commercialisation de véhicules équipés de moteurs à combustion dès 2025. Nous devons dès à présent poser un cadre chiffré, afin d'accompagner les évolutions inéluctables de la filière et d'anticiper les impacts sur l'emploi. Ainsi, les entreprises concernées par le domaine de l'automobile disposeront d'une date butoir précise,

compris aux horizons de 2023 et 2028. Les objectifs mentionnés dans l'amendement n° 800 rectifié sont cohérents avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, le contrat stratégique de la filière automobile, la feuille de route

une position centrale, qui n'est absolument pas remise en cause. Avons-nous l'intention, dans le secteur de l'automobile électrique, où la batterie représente de 45 % à 50 % du coût du véhicule, de dépendre exclusivement d'une économie centralisée, dont les moyens, nous l'avons vu pour les panneaux photovoltaïques, ne font pas appel à des principes de concurrence, sauf à désarmer nos constructeurs et à rendre les clés de la maison

établie. Enfin, quelle que soit la passion que nous ayons les uns et les autres pour l'exemplarité française, force est de reconnaître que tous les pays ne produisent pas d'électricité décarbonée comme nous le faisons, mais

encore que nous pourrons passer à travers la mutation de notre système énergétique et la sortie du thermique. Si nous ne voulons pas que ces forces,

Le scrutin est ouvert.